monsieur le ministre, mes chers collègues, Deux militaires, le premier-maître Cédric de Pierrepont et le premier-maître Alain Bertoncello, officiers mariniers au sein du commandement des opérations spéciales, ont tragiquement trouvé la mort au Sahel, au cours d'une mission ayant abouti à la libération de quatre otages, dont deux de nos compatriotes, détenus par un groupe de terroristes qui avaient sauvagement assassiné leur guide béninois. Au nom du Sénat tout entier, je tiens à saluer le courage de ces deux militaires, qui ont donné leur vie pour sauver celles des otages et à qui la Nation tout entière a rendu un hommage solennel ce matin, autour du Président de la République. Nous adressons nos pensées émues à leurs familles, à leurs proches et à leurs frères d'armes. Ce tragique dénouement nous rappelle l'engagement résolu de nos forces armées, que je tiens à saluer en votre nom à tous, pour lutter contre le terrorisme et assurer, partout dans le monde, la protection de nos concitoyens et des valeurs que nous avons en partage. Je vous invite à observer un moment de recueillement en hommage à nos deux soldats.

Mes chers collègues, le scrutin pour l'élection d'un juge titulaire et d'un juge suppléant à la Cour de justice de la République Il va être procédé, dans les conditions prévues par l'article 86 du règlement, au scrutin secret pour l'élection à la Cour de justice de la République. Ce scrutin se déroulera dans la salle des conférences, et la séance ne sera pas suspendue durant les opérations de vote. Une seule délégation de vote est admise par sénateur. Je remercie nos collègues Daniel Dubois et Annie Guillemot, secrétaires du Sénat, qui vont superviser ce scrutin. Les juges à la Cour de justice de la République nouvellement élus seront immédiatement appelés à prêter serment devant le Sénat.

du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance

Depuis un certain nombre d'années, notre école souffre de la difficulté à réduire les inégalités sociales, à permettre à tous les élèves de maîtriser les savoirs fondamentaux- lire, écrire, compter, respecter autrui -et, au-delà, à s'insérer dans la vie professionnelle.

extrémités de notre système se pose évidemment une grande interrogation sur les causes et les raisons de ces phénomènes. Bien entendu, nous avons l'impérieuse nécessité d'apporter des réponses concrètes et efficaces.

l'école primaire est la clé de l'amélioration collective de notre système scolaire et, donc, de notre Nation. Elle joue, dans l'histoire de notre République, un rôle tout particulier, un rôle emblématique : c'est par elle que tout commence pour la vie d'un enfant comme pour la République. C'est par une politique d'élévation résolue du niveau, de justice sociale et d'équité territoriale que nous pouvons hisser l'école française parmi les meilleurs systèmes au monde, ce qu'elle a su être. Nous ferons ainsi de la France, selon les voeux mêmes du Président de la République,

D'abord, la politique de l'école primaire a abouti à diviser par deux les classes de CP et de CE1 dans les territoires les plus défavorisés, permettant ainsi, au moment où je vous parle, à 190 000 élèves de bénéficier de conditions particulières pour démarrer leur vie d'élève. Cette mesure, Cette mesure, qui commence à faire ses preuves, concernera 300 000 élèves à la rentrée prochaine. Elle va évidemment de pair avec une politique pédagogique renouvelée,

mesure doit nous permettre non seulement de mener cette politique dans les territoires classés REP et REP+, mais également de consolider l'école rurale, une consolidation que le Président de la République a confirmée au cours de sa récente Il s'agit donc aujourd'hui d'une mobilisation à la fois pédagogique et budgétaire au service de l'école primaire. Le projet de loi dont nous nous apprêtons à débattre s'inscrit donc pleinement dans la priorité éducative rappelée et approfondie par le Président de la République au cours de sa conférence de presse du 25 avril il a annoncé, outre les éléments que je viens d'indiquer, la fin des fermetures d'écoles primaires sans l'accord du maire, le dédoublement des grandes sections de maternelle classées en zone d'éducation prioritaire et la limitation à 24 élèves par classe en grande section, en CP et en CE1 partout en France. Le projet de loi pour une école de la confiance s'inscrit dans une politique générale qui fait de l'éducation le coeur du projet de société que nous avons pour l'élévation du niveau général de notre peuple, mais aussi pour la justice sociale. Tant de choses ont été dites à propos de ce projet de loi

Nous pouvons avoir des points de vue différents sur chacun des articles, mais nous ne saurions décrire l'article autrement qu'il n'est. L'article 1 de ce projet de loi ne vise en aucun cas à museler les professeurs, comme je l'ai entendu. Il rappelle tout simplement à tous ceux qui ont décidé d'être fonctionnaires les droits et les devoirs afférents, qui ont été définis par des lois précédentes. Il rappelle surtout un principe essentiel sur lequel on ne peut transiger, savoir le respect de la communauté éducative par les familles. Autrement dit, non seulement cet article ne crée pas de contrainte nouvelle pour les professeurs, mais il est, au contraire, le fondement juridique d'un respect accru pour cette fonction par le reste de la société.

En cohérence avec l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, il avance l'âge de la première visite médicale à 3 ans, offrant ainsi à tous les élèves un parcours de santé entre 0 et 6 ans. Cet article, comme bien d'autres, fait de ce texte une loi profondément sociale. D'ailleurs, si je ne devais insister que sur un point, ce serait celui-là. Cette loi, qui est une loi pour l'éducation, est d'abord et avant tout une loi profondément sociale.

de transmettre. Ainsi, dès la rentrée prochaine, des étudiants en deuxième année de licence recevront 700 euros par mois, en plus de leur bourse, pour faire de l'aide aux devoirs, pour seconder les professeurs, et certainement pas pour les remplacer.

de toutes les femmes et de tous les hommes de progrès sur un tel sujet ? Pourquoi entendons-nous des propos faux en la matière, alors que nous renouons avec ce qui fait normalement consensus autour de l'école de la République ?

Il faut maintenant identifier les leviers essentiels susceptibles d'améliorer notre politique éducative et les actionner afin d'atteindre la seule chose qui compte : le progrès effectif de tous les élèves. Le premier des leviers est l'école primaire, tout particulièrement l'école maternelle. C'est là qu'il est possible d'attaquer les inégalités à la racine. Là aussi, j'ai entendu dire que le Gouvernement voulait supprimer les écoles maternelles.

à la racine. En fonction de son milieu social et culturel, un jeune enfant peut accumuler des retards linguistiques considérables. C'est pourquoi il importe tellement de faire de l'école maternelle une véritable école en abaissant l'obligation d'instruction à 3 ans. Sachez, mesdames, messieurs les sénateurs, que c'est une grande fierté pour moi d'appartenir à un gouvernement à qui le Président de la République a demandé de s'inscrire dans la lignée des grandes lois républicaines sur l'obligation scolaire. Incontestablement, il s'agit aussi évidemment

Aujourd'hui, les travaux issus de la recherche soulignent que les années passées à l'école maternelle sont décisives pour la maîtrise future des savoirs fondamentaux. Cette loi vise donc à renforcer l'école maternelle, à la reconnaître et à lui donner les moyens d'être le fer de lance de l'élévation du niveau général et de la justice sociale. L'apprentissage du vocabulaire, l'émergence progressive d'une conscience grammaticale par la lecture de livres, l'éveil de la sensibilité par les arts, le développement psychomoteur et affectif, la socialisation par le respect des règles et le jeu, le souci du travail bien fait sont des fondations indispensables pour susciter le plaisir d'aller à l'école, cette école de la confiance, une école du bonheur- j'ose ce mot -, que nous pouvons souhaiter pour tous nos enfants.

Cette hétérogénéité dans la formation n'est plus possible si l'on souhaite vraiment que tous les élèves maîtrisent les savoirs fondamentaux. Le principe d'égalité doit trouver à s'appliquer pleinement en matière de formation des professeurs. C'est pourquoi la création des Inspé est si importante. Le changement du nom indique quelque chose d'important : le « i » pour institut signifie que nous voulons fonder tout cela sur une culture professionnelle ; le « n » comme national veut dire que nous voulons un cadre commun de référence

Ce droit est la marque de confiance dans les femmes et les hommes qui travaillent au plus près des réalités et de la diversité des territoires. Libérer, protéger, unir : ces mots forment la clé de voûte de ce texte. Il n'existe pas d'expérimentation sans évaluation digne de ce nom. Ce projet de loi permet les expérimentations et les évaluations. Nous allons approfondir la culture de l'expérimentation grâce à cette loi.

en s'appuyant notamment sur l'auto-évaluation, qui est une façon de responsabiliser l'ensemble des acteurs sur leur capacité à faire progresser les élèves. En définitive, si l'école française est si consubstantielle à la République, c'est qu'elle fut, qu'elle demeure et qu'elle demeurera son visage, le visage du progrès et celui de l'avenir. Aujourd'hui, les horizons de notre école s'étendent au monde, et chacun sent bien la nécessité pour nos élèves de maîtriser parfaitement le français ainsi que des langues étrangères afin tout simplement que ceux-ci soient de leur temps et de leur espace. Aussi, nous devons développer les échanges en Europe et dans le monde. Il y va du rayonnement de la France, de sa place dans le concert des nations, de sa capacité à attirer les meilleurs talents. Actuellement, l'enseignement international est souvent réservé aux familles favorisées, celles qui peuvent scolariser leurs enfants dans des écoles privées parfois coûteuses. En soumettant à votre vote la création d'établissements publics locaux d'enseignement international, je vous propose de conférer au service public d'éducation une plus forte dimension internationale afin que les élèves venus de tous les milieux et de tous les horizons puissent bénéficier de cette dynamique et s'ouvrent encore davantage sur l'Europe et le monde.

L'école de la République, c'est la maison commune de toute la jeunesse de France. À ce titre, elle doit apporter à tous ses enfants, où qu'ils se trouvent sur le territoire, la même chance de réussir et la même envie de saisir cette chance. C'est pourquoi il revient à l'État d'assurer la protection de tous ses enfants. Si la liberté d'instruction est un droit fondamental, nous devons avoir un contrôle particulièrement vigilant sur la qualité des enseignements qu'ils reçoivent. Nous savons tous que tel n'est pas le cas partout. Ce projet de loi permet donc de renforcer cette garantie. Le texte que nous examinons est résolument un texte de confiance dans les territoires ; je le dis devant cette chambre qui a particulièrement vocation à défendre ses territoires

nous ne devons écarter aucune organisation susceptible d'aider les territoires à offrir un service d'éducation de qualité. Il revient à l'État de garantir l'équité entre les territoires, en donnant plus à ceux qui en ont besoin et en disposant d'organisations appropriées

par des moyens budgétaires supplémentaires pour accompagner cette évolution. Cette politique d'équité s'adresse particulièrement aux élèves les plus fragiles, notamment les élèves en situation de handicap. Je tiens à finir mon discours par ce point, afin de marquer qu'il s'agit, à mes yeux, d'un sujet essentiel. Beaucoup a été fait depuis le début des années 2000, avec de premières politiques importantes en la matière. le défi à relever est immense. Il nous faut changer le regard sur la différence et réussir la transformation de nos organisations. Notre ambition est claire : faire en sorte que tous les enfants dont le handicap est diagnostiqué soient pris en charge le plus rapidement possible. le levier qui vous est proposé au travers de ce projet de loi est inédit : il s'agit de faire émerger un grand service public de l'école inclusive avec 80 000 personnels mieux formés, mieux reconnus, mieux intégrés à l'équipe éducative, répartis sur tout le territoire en pôles, et qui, en toutes circonstances, sur le temps scolaire et périscolaire, accompagneront les enfants en situation de handicap. Nous voulons que, dès la rentrée prochaine, cette amélioration soit visible pour les élèves et leurs familles, ainsi que pour les personnels accompagnants.

la rentrée, que l'organisation des établissements soit de nature à assurer un accompagnement au plus près des besoins des élèves. Nous voulons avoir une approche qualitative complémentaire de l'approche quantitative, pour que les accompagnants se sentent membres à part entière de la communauté éducative.

donner un socle à cette espérance dont nous avons besoin et dont nous nous donnons maintenant les moyens. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi porte une ambition : permettre à l'école de demeurer l'institution par laquelle tout est possible. Cela a été dit à plusieurs reprises par le Président de la République, le Premier ministre et moi-même. Nous pouvons considérer l'école comme le premier des outils dont nous disposons pour la justice sociale. Pour ce faire, il est nécessaire de repenser le lien de l'école avec les familles, en accueillant mieux les enfants en situation de handicap et en posant comme fondement de cette relation l'esprit de confiance. Cette école de la confiance que nous appelons de nos voeux est non pas un mot, mais une aspiration sociale profonde conduisant à plus de liberté, plus d'unité et aussi plus de protection. Nous évoluons beaucoup trop dans une société de défiance ; tel est le diagnostic que nous pouvons faire sur notre pays. Or ce diagnostic date non pas d'hier, mais de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Il n'a pas toujours caractérisé la société française. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir de nouveaux leviers pour créer un cercle vertueux de la confiance. À cet effet, une loi ou un décret ne suffit pas. Il nous faut enclencher le cercle vertueux de la confiance

! ... et en tenant compte des amendements- c'est ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale et c'est ce que je ferai au Sénat. Nous sommes sauvés ! C'est pourquoi se trouve au coeur de ce projet de loi une philosophie de la confiance, qui converge avec une philosophie de la démocratie parlementaire.

Notre démarche consiste à placer au centre de l'école les professeurs, sans lesquels rien n'est possible. Mieux les aider pour entrer dans le métier, leur offrir une formation de qualité, faire respecter leur autorité, tel est mon devoir et tel est mon objectif avec ce projet de loi. Mesdames, messieurs les sénateurs, je suis fier de vous présenter un texte de nature à permettre à la France de porter une politique éducative ambitieuse. Par ce projet, nous souhaitons donner à nos enfants des racines et des ailes Oh là là ! ... la fierté d'être des citoyens de France, la fierté d'être eux-mêmes.

mais nous avons surtout cherché à l'améliorer, à le compléter, à le densifier. Et si notre regard a été critique, peut-on d'ailleurs nous le reprocher ? regard a été critique, parce que nous avons dit que ce texte péchait par sa méthode d'élaboration, une méthode faisant trop souvent fi de la concertation et du dialogue social, ainsi que l'illustrent l'introduction à l'Assemblée nationale des établissements publics locaux des savoirs fondamentaux, un chapitre entier sur l'école inclusive ou encore les multiples habilitations à légiférer par voie d'ordonnance. regard a été critique, parce que nous avons aussi indiqué que, à l'aune de l'ambition d'une élévation générale du niveau des connaissances, d'une école plus juste, qui aurait retrouvé la confiance de la société et et confiance en la société, ce projet de loi était incomplet par son contenu. Certes, en abaissant l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans, votre projet de loi prévoit une avancée démocratique que l'école n'avait pas connue depuis les lois fondatrices de Jules Ferry. Mais, reconnaissons-le ensemble, ce progrès demeure symbolique, puisqu'il ne concernera, dans les faits, que 2 % à peine des enfants d'une classe d'âge, les autres ayant déjà rejoint, par la volonté des parents, les bancs de l'école maternelle. La mesure emblématique, qui est la raison d'être de ce projet de loi, est donc, pour l'essentiel, une mesure d'adaptation. Hormis en Guyane et à Mayotte de celle-ci se heurtera à de grandes difficultés, cette disposition se révélera sans réel impact sur les autres territoires français. En l'espèce, la loi ne fait que suivre le mouvement que la société a déjà imprimé. Quant aux autres dispositions, elles sont d'importance très variée, alors qu'un volet demeure absent, celui des mesures relatives à la gestion des ressources humaines et aux conditions d'exercice du métier d'enseignant. Il s'agit pourtant là du levier majeur d'amélioration de notre école. Comme les événements récents en témoignent, il est de plus en plus évident que les professeurs n'ont plus confiance en leur hiérarchie et ne se sentent plus ni écoutés ni considérés. Or la valeur de l'école se mesure aussi à l'aune du moral de ses professeurs. Puisqu'il devait finalement y avoir une loi, alors, oui, l'école de la République, notre école, méritait plus. Car il y a urgence. Les évaluations se succèdent et les acquis des élèves qu'elles mesurent se dégradent. L'échec scolaire se caractérise par sa précocité croissante et l'incapacité de notre système éducatif à le réduire. Il a raison ! Plus grave, la promesse républicaine fondatrice de notre école régresse. Notre système éducatif devient à l'opposé de cette promesse : il est l'un des plus inégalitaires des pays développés. Ses faiblesses, monsieur le ministre, vous les connaissez, et vos actions sont tendues vers leur résolution. Si la perspective dans laquelle s'est inscrite la commission était donc résolument et raisonnablement critique, elle est tout aussi résolument et raisonnablement constructive. En effet, mes chers collègues, votre commission a souhaité demeurer fidèle à ce qui fait l'intérêt du Sénat : un attachement à la qualité de la loi, en rejetant les dispositions bavardes, superflues ou manifestement réglementaires ; un esprit d'ouverture et de compromis une attitude pragmatique et la prise en compte de la diversité des réalités locales. Votre commission a aussi cherché à dépasser les clivages pour avoir un débat de qualité, un débat digne de l'école, parce que notre école le mérite

Le texte adopté par la commission est le fruit de ce travail collectif, dont je suis particulièrement fier : 141 amendements de presque tous les groupes ont permis de construire un texte plus équilibré et plus abouti, portant la voix des territoires jusqu'alors trop négligée. La commission a ainsi apporté de nombreuses améliorations au texte qui lui était soumis. Elle a réécrit l'article 1 pour rappeler que l'exigence d'exemplarité est au service de l'autorité des professeurs et pour réaffirmer une relation d'autorité dans laquelle le respect est d'abord et avant tout dû par les élèves et leurs familles aux personnels et à l'institution scolaire. S'agissant de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, votre commission n'a pas remis en cause cette mesure, mais elle a été attentive aux conditions de son application. Elle a veillé à donner de la liberté aux parents, en pérennisant la dérogation permettant aux jardins d'enfants d'accueillir des enfants de 3 à 6 ans. Elle a souhaité donner de la souplesse, en formulant des dérogations à l'obligation d'assiduité. Enfin, elle a modifié l'article 4 pour assurer la juste compensation des communes qui soutenaient déjà les écoles maternelles privées sous contrat. À l'article 5, elle a souhaité donner aux familles les garanties d'un contrôle équitable, sans pour autant nuire à l'effectivité de ce dernier. Elle a renforcé substantiellement le volet consacré à l'école inclusive, visant notamment à créer les modalités d'un accompagnement de qualité et à améliorer les conditions de travail et de formation des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Se faisant l'écho de l'incompréhension suscitée par l'article 6 , votre commission l'a supprimé, afin d'envoyer un signal fort au Gouvernement et au pays. Nous examinerons lors de nos débats un amendement de notre collègue Jacques Grosperrin tendant à rétablir cet article en donnant de solides garanties aux élus locaux, aux enseignants, aux directeurs et aux parents. Notre commission a approuvé le principe de l'évaluation des établissements et de l'instauration du conseil d'évaluation de l'école à l'article 9. Elle a toutefois revu la composition de l'instance, afin d'en renforcer l'indépendance vis-à-vis du ministre et du Gouvernement. Elle a ainsi prévu la nomination de son président par le chef de l'État et renvoyé la nomination des six personnalités qualifiées aux présidents des assemblées parlementaires et au Premier ministre. Elle a fixé à six ans la durée de leur mandat, afin que celui-ci dépasse les alternances politiques. Notre commission a travaillé enfin à combler les lacunes de ce texte, en introduisant plusieurs dispositifs de gestion des ressources humaines qui font aujourd'hui défaut la poursuite des actions de formation initiale au cours des trois premières années de carrière ; l'obligation de formation continue pour tous les enseignants, organisée prioritairement en dehors des heures de classe ; les premiers jalons d'un statut du directeur d'école ; l'association du chef d'établissement aux décisions d'affectation qui concernent son établissement, mais également la création d'un contrat de mission permettant d'affecter dans les établissements les plus difficiles des enseignants chevronnés et motivés. Enfin, la commission a supprimé l'article 17, considérant qu'un blanc-seing ne pouvait être donné à une mesure aussi importante pour nos territoires que l'organisation des rectorats. Je constate avec satisfaction que le Gouvernement a joué le jeu et proposé d'inscrire dans la loi les dispositions de l'ordonnance prévue. Vous le voyez, mes chers collègues,

seront l'occasion de continuer d'enrichir ce projet de loi dans l'intérêt de l'école et de la réussite des élèves de ce pays ! Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'espère que nous aurons un débat digne de notre école.

L'école n'a pas besoin, à chaque alternance politique, d'une nouvelle loi. Elle peut se gouverner autrement. » Vous avez tenu parole. en peu de temps, sans recourir à la procédure législative, vous avez profondément modifié l'organisation, les finalités et le fonctionnement de l'éducation nationale, en transformant considérablement l'enseignement professionnel, le baccalauréat, le lycée et les programmes. De toutes ces réformes, la Haute Assemblée n'a pas eu à connaître, hormis dans le cadre des débats qu'elle a elle-même convoqués. Très récemment, M. Pierre Mathiot déclarait à propos de la réforme du baccalauréat : « C'est C'est une réforme qui est lourde, structurelle, et qui concerne un secteur qui n'a pas été réformé depuis un demi-siècle. » Il eût été légitime que le Sénat vous entendît sur les finalités d'un changement aussi radical. À ces bouleversements majeurs s'ajoutent les restrictions considérables imposées à l'accès à l'enseignement supérieur par la loi relative à l'orientation et la réussite des étudiants, que votre collègue continue de nous présenter comme une remédiation strictement technique au recours illégal au tirage au sort. Progressivement, parents et enseignants comprennent que toutes ces réformes font système et que, loin d'être dictées par des nécessités pratiques, elles sont inspirées par une pensée politique globale, que vous n'assumez pas. Parents et enseignants mesurent, de plus en plus, le décalage profond qui existe entre les déclarations officielles et la réalité telle qu'ils l'éprouvent dans les établissements. Cette distorsion entretient du doute, de l'inquiétude et, finalement, de la suspicion. Élus de terrain, nous avons mesuré, ces dernières semaines, combien la défiance était grande envers des mesures dont nos concitoyens perçoivent qu'elles sont dictées par des objectifs dont on leur cache le dessein essentiel. Vous avez parlé de « bobards », monsieur le ministre ; nous percevons surtout de l'incompréhension, du soupçon et de la méfiance. La loi que vous nous proposez aujourd'hui aurait pu être l'occasion d'une déclaration clarificatrice sur vos intentions politiques véritables. La commission de la culture du Sénat a considéré qu'elle était, tout au contraire, bavarde, peu lisible et confuse. Je partage sur ces points les critiques exprimées à l'instant par notre rapporteur, le sénateur Max Brisson. L'objet de cette loi était de rétablir la confiance entre le corps enseignant, son ministère de tutelle et les parents. Je crains qu'elle n'entretienne davantage la défiance. Enfin, et surtout, alors que nous dressons le constat commun d'une école incapable de corriger les inégalités sociales d'accès au savoir, votre projet est dépourvu de l'ambition de mobiliser les ressources de la Nation pour rebâtir une éducation nationale au service de l'émancipation, du développement humain et de l'égalité des droits politiques. Nous aurions pu, ensemble, réaliser pour le XXI siècle la généreuse utopie que Condorcet esquissait ainsi en 1792, « an IV de la liberté » : « Assurer [à tous les individus de l'espèce humaine] la facilité de perfectionner son industrie, de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a droit d'être appelé, de développer toute l'étendue des talents qu'il a reçus de la nature ; et par là, établir entre les citoyens une égalité de fait, et rendre réelle l'égalité politique reconnue par la loi. Nonobstant certaines dispositions qui auraient pu être mises en oeuvre par la voie réglementaire, l'objet législatif principal de ce texte est de satisfaire l'annonce présidentielle de l'abaissement de l'âge de la scolarisation obligatoire à 3 ans. Et encore, les maires ont vite compris qu'elle se réaliserait grâce à la contribution des finances municipales. Historiquement, cette loi apparaît alors comme l'extension, jusqu'à cet âge, des mesures pécuniaires de la loi du 31 décembre 1959, dite loi Debré. Toutefois, son manque d'ambition l'en distingue absolument. La loi Debré portait à 16 ans la scolarité obligatoire. Cette extension s'accompagna d'un programme massif de recrutement d'enseignants. Dans le même temps, de 1960 à 1969, la taille moyenne des classes des écoles primaires publiques fut réduite de 30 à 26 élèves, ce qui imposa l'embauche de 4 000 instituteurs pendant ces dix années. Alors que la dépense publique est aujourd'hui considérée comme un abject vice par la doxa libérale, Louis Cros, haut fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale, expliquait ainsi, en 1961, les nécessités d'un investissement massif de l'État gaullien dans l'enseignement : « Pour la première fois dans l'histoire, les aspirations idéalistes et les nécessités pratiques en matière d'enseignement ont cessé de se contredire. En France, les exigences de la prospérité et de l'équilibre économique s'ajoutent maintenant aux raisons de justice et d'égalité sociale pour rendre nécessaire, en même temps que désirable, l'instruction la plus développée possible pour le plus grand nombre possible d'enfants. La France a besoin de développer toutes ses ressources intellectuelles. Sinon elle deviendrait un pays intellectuellement sous-développé, qui maintiendrait artificiellement une économie anachronique à coup de subventions économiques, ou d'indemnités de chômage quand des générations plus nombreuses parviendront à l'âge d'homme. » Brillante prophétie ... Près de soixante ans plus tard, nous pourrions dresser le même constat et nourrir la même ambition. L'accélération du progrès technique, la révolution du numérique et la quantité exponentielle d'informations que nous devons traiter tous les jours exigeraient sans nul doute que notre enseignement franchisse une nouvelle étape. Ne serait-il pas temps, par exemple, de prolonger l'enseignement obligatoire jusqu'à la majorité ? C'était l'une des préconisations du plan conçu, à la Libération, conformément au programme de gouvernement du Conseil national de la Résistance, par Paul Langevin et Henri Wallon. Combien de temps nous faudra-t-il encore pour réaliser cette élévation supplémentaire de la durée d'instruction ou de formation pour celles et ceux qui, trop nombreux, la quittent toujours, sans diplôme, à 16 ans ? Certes, votre projet instaure une obligation de formation pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans, mais, comme l'a montré notre commission, cette mesure est symbolique. L'abaissement de l'âge de la scolarisation à 3 ans l'est tout autant en France métropolitaine. Il demandera toutefois un véritable effort pour être appliqué dans les outre-mer et, sur ce point, nous attendons de votre gouvernement des engagements fermes et précis. En substance, ce qui caractérise ce texte, c'est son manque d'ambition pour l'école. L'accumulation de mesures techniques, souvent discutables, ne peut cacher cette vacuité. Elle est d'autant plus décevante que, dans le même temps, selon la formule consacrée, le Président de la République annonçait, le 25 avril dernier, un plan d'investissement massif en faveur de l'école. Les promesses donnent le vertige dédoublement de 6 000 classes supplémentaires, limitation à 24 du nombre d'élèves dans toutes les classes de la grande section de maternelle au CE1, revalorisation du métier de professeur, moratoire pour la fermeture des classes, etc. Pour assurer seulement le dédoublement des classes, dans son programme, le candidat Emmanuel Macron avait estimé à 12 000 postes le besoin de recrutement. Nous ne doutons pas de la volonté du Président de la République d'honorer rapidement ses engagements. Votre collègue en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche a lancé une grande concertation dont les conclusions fourniront la matière d'une grande loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui sera présentée au Parlement avant la fin de l'année. Pour satisfaire les ambitions du Président de la République en faveur de l'école, nous vous proposons la même méthode. C'est l'objet de cette motion tendant à opposer la question préalable : nous donner collectivement le temps de préparer ensemble, avec tous les acteurs de l'éducation, la grande loi dont l'école de la République a besoin, pour, selon les mots de Condorcet, « contribuer contribuer [au] perfectionnement général et graduel de l'espèce humaine, dernier but vers lequel toute institution sociale doit être dirigée ». La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre groupe s'opposera à cette motion tendant à opposer la question préalable, déposée par le groupe CRCE. Certes, nous avons noté les faiblesses du projet de loi, pour ne pas dire son absence de contenu. Vous aviez d'ailleurs déclaré, au début de votre mandat, monsieur le ministre, qu'il n'y aurait pas de « loi Blanquer », car vous-même n'en ressentiez pas la nécessité. Le Gouvernement a surtout fait un acte de communication en affichant plusieurs messages symboliques. Tout d'abord, la mesure phare du projet de loi, l'abaissement à 3 ans de l'instruction obligatoire. Celle-ci ne concernera pourtant qu'une infime proportion d'enfants, beaucoup étant déjà scolarisés dès 3 ans. De même, la confiance prônée par le projet de loi est censée s'appuyer sur un respect mutuel, qu'il est aisé de décréter. Quant au principe d'une formation obligatoire entre 16 et 18 ans, c'est une sorte de voeu pieux, qui ne règle en rien le problème crucial de la déscolarisation. Le reste du projet de loi permet d'adopter diverses mesures d'intérêt varié et sans grande cohérence. Nous partageons donc le sentiment d'un manque d'ambition du texte. Cependant, le projet de loi a été remanié en commission. Notre rapporteur Max Brisson, dont je salue la qualité du travail, s'est attaché à corriger les défauts et les oublis du texte. Ainsi, plutôt que de les placer sur un même plan, la commission a rappelé la place majeure de l'autorité de l'enseignant sur les élèves. Elle a introduit de la souplesse dans l'application du principe de scolarisation à 3 ans et garanti la compensation pour toutes les communes concernées. Elle a complété le chapitre dédié à l'école inclusive pour un meilleur accompagnement des élèves en situation de handicap. Elle a rassuré parents, enseignants, directeurs et élus locaux, en supprimant l'article 6 , qui a fait grand bruit en étant introduit sans concertation préalable à l'Assemblée nationale. La commission a également traité de sujets qui ne figuraient pas dans le projet de loi, mais sur lesquels nous appelons à légiférer de longue date, comme le statut des directeurs d'établissements ou la formation continue. Je n'irai pas plus loin, car la liste est longue : quelque 141 amendements ont été adoptés en commission pour redessiner le texte. Notre groupe estime dès lors qu'il serait regrettable d'effacer et d'interrompre ce travail sénatorial, en renvoyant ainsi un texte inachevé et bancal aux députés. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette motion. Quel

subtilité avec laquelle vous avez analysé la question de la loi, au début de votre intervention. Il est exact que le sujet de l'éducation relève d'une hiérarchie des normes particulière, qui ne dépend pas de moi et qui mérite d'être discutée.

pas de vous offusquer si, demain, des députés me reprochaient d'avoir pris en compte des amendements sénatoriaux. Je prendrai évidemment en compte tous les amendements au cours de cette discussion,

la démarche de nos collègues du CRCE, mais le groupe La République En Marche votera contre la motion tendant

est à M. Stéphane Ravier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte aurait dû être fondamental, mais il est au final bien décevant : aucun cap, aucune vision, aucun changement, même pas de « nouveau monde » ... On y retrouve toutes les dérives de ce monde de déracinés porté par les idéologues du ministère de l'éducation nationale depuis des années. On remplace les termes « intégration dans la société » par « société inclusive » : c'est tout le symbole de la disparition d'une vision globale de la communauté, du bien commun et de la Nation.

Cette confiance, elle se mérite et se gagne en créant les conditions favorables à son éclosion, et ces conditions ne sont en rien réunies dans ce texte. Il faut en réalité changer totalement de cap, en redonnant du sens à l'autorité du professeur sur les élèves. L'élève ne saurait être l'égal du maître. Le maître est là pour enseigner, pour transmettre ; l'élève pour écouter, apprendre, comprendre dans le respect absolu de son professeur. On se souvient tous de cette vidéo d'un professeur braqué par un élève avec une arme qui s'est révélée être factice, et de toute la polémique du hashtag #PasDeVague d'un corps professoral qui n'en peut plus de cette violence devenue quotidienne. Rien donc sur l'insécurité à l'école ! Vous préférez au contraire rappeler le devoir de réserve des professeurs dès l'article 1. « Ouvrez une école, et vous fermerez une prison », disait en son temps Victor Hugo. Aujourd'hui, ce sont les professeurs qui sont incarcérés dans leur classe, isolés derrière les barreaux de la violence issue des quartiers ethniques et de l'indifférence de leur ministre de tutelle Rien sur les programmes désastreux qui nous font plonger chaque année plus bas dans le classement PISA ; rien sur le poids de l'immigration, ... Il y avait longtemps ! ... qui, de toute évidence, constitue, là aussi, un véritable fardeau, contribuant à l'effondrement du niveau scolaire À croire que, demain, quand cette loi sera votée, les classes en ruralité pourront continuer de disparaître, et les établissements de REP et REP+ continuer de péricliter. Quant aux élus locaux, ils seront plus abandonnés encore dans la gestion des établissements. De plus, ce regroupement des écoles et des collèges en établissements publics de savoirs fondamentaux s'apparente à la création d'une superstructure qui compliquera davantage la tâche des élus locaux. Il supprime la présence de l'interlocuteur primordial pour les parents d'élèves qu'est le directeur d'école et constitue la menace de voir à terme la suppression de postes et d'écoles. On ajoute à cela l'apparition des termes « parent 1 » et «parent 2 » dans les formulaires scolaires, une véritable provocation qui ne semble pas heurter la majorité de droite du Sénat, et qui est tellement révélatrice de la place qu'occupe l'idéologie dans nos institutions, y compris, et même surtout, au sein de l'institution scolaire. Finalement, l'instruction obligatoire à 3 ans représente une nouvelle contrainte pour les familles et les collectivités locales. C'est en réalité un pur gadget pour faire croire que tout change, alors que rien ne change. Les bases essentielles nécessaires au savoir, qui permet à chaque enfant devenu adulte d'être libre,

l'examen du projet de loi pour une école de la confiance, que nous entamons aujourd'hui, marque l'aboutissement d'un intense travail préparatoire. Je tiens à remercier dès à présent notre collègue rapporteur, Max Brisson,

nous avons tous été saisis ou alertés à propos de telle ou telle disposition du texte qui pouvait inquiéter. Le déchaînement des passions qu'entraîne bien souvent un projet de loi sur l'éducation nationale

évidence. Il trouve son origine dans la volonté du Gouvernement de généraliser l'instruction des enfants dès l'âge de 3 ans. Si cette mesure ne concerne, en métropole, que quelques milliers d'enfants, elle est cependant motivée par un objectif, que nous partageons, d'égalité scolaire et sociale, et de détection précoce des maladies ou situations de handicap.

Des craintes ont pu être exprimées quant à une mainmise plus importante du ministère sur ce nouvel organisme, ce à quoi notre commission a, là encore, apporté une réponse qui saura, je l'espère, satisfaire

Au-delà de ces problématiques purement scolaires, le texte contient une série de dispositions appelant, notamment, à une meilleure prise en compte du handicap dans l'école et autour d'elle, à une revalorisation du statut des accompagnants, ainsi qu'à des mesures de sensibilisation destinées aux élèves.

À ce sujet, le texte prévoit notamment la création des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les PIAL. Ce dispositif vise à coordonner, au sein des établissements scolaires, les moyens humains dédiés à l'accompagnement des élèves en situation de handicap.

n'a pas forcément été facile. Le rapport de Pierre Mathiot et Ariane Azéma, devait être présenté en juin ; il aurait pu calmer les tensions et nourrir la réflexion sur ce sujet, mais la manière dont a été inséré cet article n'a fait qu'aviver les craintes et les crispations.

dépôt du projet de loi et qui, bien entendu, en modifient certains aspects. Je tiens à le souligner, le groupe des sénateurs centristes entend néanmoins proposer une réponse aux craintes concernant des fermetures de classe. Enfin, le texte prévoit le recours à l'expérimentation pour les établissements, dans un cadre défini et contrôlé. Ce droit à l'expérimentation nous semble nécessaire pour permettre à l'éducation d'évoluer et de s'adapter aux nouveaux besoins pédagogiques et territoriaux il pourrait toutefois être plus ambitieux et concerner des champs plus larges, notamment sur le plan administratif. C'est en effet une conviction que nous portons : dans le domaine de l'éducation nationale, où la moindre évolution

Le projet de loi pourrait aller plus loin en la matière ; tel est le sens d'amendements que nous défendrons. Si le texte pouvait redonner confiance aux acteurs locaux pour prendre des initiatives, alors, dans ce cas, le nom donné au projet de loi prendrait certainement de sens. Mes chers collègues, voici le résultat du scrutin pour l'élection d'un juge titulaire et d'un juge suppléant à la Cour de justice de la République Nombre de votants : 271 Suffrages exprimés : 242 Majorité absolue des suffrages exprimés : 122

; Mme Muriel Jourda, suppléante, 242 voix. Ces candidates ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, elles sont proclamées juges à la Cour de justice de la République. la République vont être appelées à prêter, devant le Sénat, le serment prévu par l'article 2 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. » Acte est donné par le

Acte est donné par le Sénat du serment qui vient d'être prêté devant lui. Nous

Cette évolution, qui s'impose à nous, nous invite à inventer le monde de demain ; vaste entreprise ! Aussi, monsieur le ministre, lorsque vous avez présenté votre vision de l'école de demain-

Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui a donc vocation à s'inscrire parmi les grandes lois républicaines sur l'école qui ont marqué notre temps. En 1882, la loi Ferry instaurait l'âge obligatoire d'instruction à 6 ans en 1936, près de cent ans après l'adoption des premières lois sur l'interdiction du travail des enfants, l'école était rendue obligatoire jusqu'à 14 ans ; puis, en 1959, elle le fut jusqu'à 16 ans. En 2019, le Gouvernement souhaite, en même temps, abaisser l'âge obligatoire de la scolarité à 3 ans et proposer une obligation de formation ou d'activité pour les jeunes de 16 à 18 ans.

de transformer une liberté d'instruction précoce, déjà largement diffusée en France, en obligation légale. Ce qui est présenté comme le fer de lance de l'État contre la reproduction des inégalités sociales et la lutte contre l'échec scolaire ne concernera que 26 000 enfants par classe d'âge, tandis que l'échec scolaire concerne plus de 100 000 élèves par an ... Au grand dam des élus locaux, le projet de loi initial ne prévoyait pas de pleine compensation des charges occasionnées pour les communes,

Nous nous félicitons des aménagements d'assiduité prévus dans le cadre de la première année d'école maternelle, adoptés lors de l'examen du texte en commission. La France présente une particularité : celle d'une école qui s'administre de façon collégiale, quand le système éducatif est, partout ailleurs, étroitement hiérarchisé. Cette question suscite des débats depuis bien longtemps, depuis l'apparition des établissements publics de l'enseignement primaire, institués par François Fillon. Depuis lors, les rapports se sont multipliés et la question reste posée Notre commission de la culture a introduit une mesure instaurant un lien hiérarchique entre le directeur d'école et les professeurs. En réalité, les directeurs d'école ont besoin d'une évolution pour mieux gérer leur école ; surtout, il serait temps de créer, dans le cadre d'une

La première finalité de l'école est de permettre à chaque élève de trouver un métier, une place dans la société, correspondant dans la mesure du possible à ses aspirations individuelles. Plus d'efforts, plus d'argent investi aujourd'hui dans notre système éducatif, c'est moins de chômage, moins de misère dans le monde de demain. Aussi, nous devons tout mettre en oeuvre pour améliorer la qualité de l'enseignement, les conditions de travail des enseignants et favoriser la réussite des élèves. Après l'acquisition des savoirs fondamentaux, la maîtrise des langues étrangères est un autre cheval de bataille pour la France ; vous l'avez souligné, monsieur le ministre. La diffusion des établissements publics locaux internationaux est un levier intéressant pour renforcer l'ouverture de notre système éducatif à l'international. La deuxième finalité de l'école est de forger chez chacun un certain sens de la citoyenneté, en proposant un terreau de valeurs, celles qu'incarne la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi de développer le sens critique, pour que chacun puisse exercer ses devoirs au sein de la société en toute indépendance d'esprit, sans tomber dans le piège de la désinformation, qui sclérose notre démocratie. Enfin, il nous appartient, au travers du réseau d'écoles, de collèges et de lycées qui maille notre territoire, de sensibiliser les élèves dès le plus jeune âge aux grands défis du XXI siècle : la préservation de l'environnement et la protection du modèle démocratique. est le sens de certains des amendements que notre groupe défendra. Monsieur le ministre, le groupe Les Indépendants - République et Territoires ne croit pas à un grand soir de l'éducation qui bouleverserait en totalité le système, et qui risquerait de casser ce qui marche sans remédier à tous ses défauts.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de commencer mon propos, permettez-moi d'adresser un message de soutien et de solidarité aux familles et à la communauté éducative du collège Gran Man Difou de Maripasoula en Guyane, endeuillées par le suicide d'une jeune aide-documentaliste. Ce drame nous rappelle douloureusement le phénomène insupportable des suicides, qui touche depuis trop longtemps nos concitoyens amérindiens et contre lequel l'école a sans nul doute un rôle fondamental à jouer. Nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder l'examen d'un texte important pour la République. Le projet de loi pour une école de la confiance est en effet un marqueur de la politique engagée par le Gouvernement en faveur d'une « élévation du niveau général des élèves » et d'une école plus juste. Dégradation des performances et des acquis, décrochage scolaire et inégalités : notre école doit relever de nombreux défis. Ce texte ne saurait, à lui seul, y répondre, parce que tout ne relève pas de la loi, mais aussi parce qu'il s'inscrit avec cohérence dans une politique bien plus ambitieuse. Il est vrai que, depuis son adoption à l'Assemblée nationale, de vives inquiétudes ont été exprimées, parfois en raison d'imprécisions réelles, le plus souvent à cause de rumeurs et de contre-vérités, qui touchent les fondements mêmes de la démocratie. Monsieur le ministre, vous avez engagé un dialogue essentiel avec les principaux acteurs et rassuré quant à votre volonté d'améliorer ce projet de loi, afin, vous l'avez souvent répété, qu'il soit mieux compris par chacun. Le dialogue va se poursuivre dans cet hémicycle ; en tout cas, je l'espère. Cela nous permettra d'apporter les clarifications nécessaires et de faire la lumière sur les véritables mesures proposées. « Incohérent », « symbolique », voire « inutile » ; beaucoup de choses ont été reprochées à ce texte, en oubliant parfois sa portée éminemment sociale. Social, ce

Il est vrai que, avec 98 % d'enfants de 3 ans déjà scolarisés, cette mesure accompagne un mouvement déjà imprimé par la société ; mais il est aussi vrai que, derrière les 2 % restants, se cachent d'immenses inégalités sociales et territoriales. Ce simple état de fait devrait convaincre chacun d'entre nous de la nécessité de légiférer, pour faire en sorte que la promesse républicaine soit tenue pour tous les Français. Dans le détail, ce sont plus de 25 000 enfants supplémentaires qui rejoindront les bancs de la maternelle à la rentrée prochaine,

Je préfère le dire, malgré l'engagement réel de l'État, les communes guyanaises et mahoraises ne seront pas en mesure d'accueillir, faute de places, tous les enfants en septembre prochain. Les expériences de double vacation sont une première réponse, mais ce n'est pas suffisant. À titre d'exemple, il faudrait construire une nouvelle école tous les neuf mois dans une ville comme Saint-Laurent-du-Maroni pour répondre à la pression démographique. Il nous faut donc donner plus de souplesse aux élus dans la construction d'infrastructures. Notre rapporteur l'a bien compris, et je tiens à l'en remercier. l'est encore lorsqu'il propose d'instaurer une obligation de formation pour tous les jeunes de 16 à 18 ans, l'objectif étant que, à l'horizon de 2020, aucun jeune ne soit dépourvu d'un emploi ou d'une formation. la mesure où il renforce, avec le prérecrutement, l'attractivité du métier de professeur, pour en faire ce qu'il a toujours été : une voie de promotion sociale. loi l'est enfin, en ce qu'il renforce l'école inclusive. Nous le savons, c'est une révolution que nous devons engager. Je pense aux accompagnants d'élèves en situation de handicap, qui doivent être considérés comme de véritables membres du personnel de l'éducation nationale. Je pense également aux pôles inclusifs d'accompagnement localisés, qui permettront d'avoir une approche au plus près des élèves, y compris par le biais du personnel médico-social. Enfin, dans le prolongement de ces mesures, le projet de loi instaure de nouveaux outils pour les territoires. C'est le cas avec la création d'un rectorat de plein exercice à Mayotte et la réforme des instances locales C'est aussi le cas avec la création d'établissements publics locaux d'enseignement international, les EPLEI, et d'établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux, les EPLESF, sur lesquels je reviendrai. Avant l'examen en séance, je veux saluer le travail de notre commission,

l'exemplarité. Notre commission a réécrit l'article 1 en conservant cette notion, qui nous semble essentielle. Toutes les disciplines scolaires ont en elles-mêmes des vertus éducatives, et, dans les yeux d'un enfant, tout adulte est un éducateur potentiel. À cet égard, loin d'être un instrument pour museler les enseignants, cet article rappelle ce qui fonde la relation entre le maître et l'élève. Deuxième principe : la libre administration des collectivités territoriales. C'est à ce titre que certaines communes avaient fait le choix de participer à la prise en charge partielle des dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées,

Si nous sommes naturellement favorables à un statut, nous rappelons que ce lien hiérarchique est loin de faire l'unanimité parmi les directeurs eux-mêmes. C'est pourquoi il semble essentiel que ce statut soit le fruit d'un dialogue avec les syndicats. enfin : l'innovation territoriale. Notre commission a envoyé un signal fort en supprimant l'article 6 , qui crée les EPLESF. Nous espérons néanmoins pouvoir en débattre à nouveau dans les prochains jours, afin de trouver une rédaction qui rassure tous les acteurs. Ces établissements doivent rester un outil, une innovation pour les territoires qui en expriment le besoin, et non une menace pour l'ensemble du système éducatif. Mes chers collègues- les nombreuses sollicitations dont nous avons fait l'objet dans nos territoires et un peu partout en témoignent -, les Français attendent du Sénat qu'il clarifie la situation. Gageons que nous serons à la hauteur, dans l'intérêt de tous nos enfants. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, même après vous avoir écouté très attentivement, monsieur le ministre, je trouve toujours aussi curieux d'avoir intitulé ce texte « projet de loi pour une école de la confiance Une école de la confiance conforterait le lien étroit, le lien de confiance, précisément, entre la commune et l'école, ces deux piliers de la République, auxquels nos concitoyens sont d'autant plus attachés qu'ils se sentent abandonnés, la plupart des services publics disparaissant dans bien des territoires. Or vous tentez de briser ce lien, d'accélérer les regroupements, de créer des établissements « XXL », éloignés, avec des chefs d'établissement missionnés plutôt pour gérer des moyens financiers et des ressources humaines que pour enseigner. Nous nous réjouissons que, lors de son passage en commission, au Sénat, votre projet se soit délesté des établissements publics des savoirs fondamentaux, qui suscitent tant de méfiance de la part des parents d'élèves, des enseignants et des élus locaux. Cette méfiance est née de l'expérience, car ces élus voient en effet se multiplier, sur le terrain, les appels à considérer l'échelon intercommunal comme la nouvelle maille de l'organisation scolaire.

Il serait regrettable que le Sénat, la chambre des territoires, soit sourd à ce qu'ils expriment et fasse entrer par la fenêtre ce qui vient d'être sorti par la porte, avec des conséquences évidentes pour le maillage scolaire, en particulier dans les territoires ruraux. Une école de la confiance viserait la réduction des inégalités sociales, territoriales et scolaires, qui, bien souvent, se confondent, en ambitionnant la réussite de tous, tout particulièrement dans un moment où grondent, en France, une colère très grande et une exigence tout aussi grande de justice sociale. Or la création des établissements publics locaux d'enseignement international, où seraient dispensés, durant toute la scolarité, des enseignements en français et en langue vivante et dont le budget pourrait comprendre des dons privés, nous semble clairement tourner le dos à cet objectif.

Une école de la confiance accompagnerait les communes dans la mise en oeuvre de l'instruction obligatoire dès 3 ans, pour en faire un élément de progrès partagé.

pourrait, en parallèle, étendre l'obligation de la scolarisation à 18 ans, comme nous le proposions au travers d'un amendement, qui a malheureusement été déclaré irrecevable. Ce serait une bien meilleure manière de lutter contre le décrochage que l'obligation de formation

Une école de la confiance se donnerait aussi les moyens d'être enfin à la hauteur de la loi de 2005 pour l'inclusion des enfants handicapés, en assurant la formation de leurs accompagnants, en dotant ceux-ci d'un véritable statut et en leur garantissant un salaire décent, afin de sécuriser et d'anticiper l'accueil des enfants. On sait combien les rentrées sont de plus en plus chaotiques La mutualisation des accompagnants, synonyme de réduction des moyens, constitue l'exact opposé de ces mesures nécessaires et nous éloigne d'une école véritablement inclusive. Une école de la confiance se fierait à ceux qui l'incarnent et la font vivre au quotidien, je veux bien entendu parler des enseignants, qui, certes, ont des obligations, conformément à leur mission de fonctionnaires, mais qui n'en restent pas moins des citoyens et des formateurs de futurs citoyens. Leur interdire la moindre critique publique à l'encontre des choix politiques de leur ministère de tutelle n'est pas une bonne chose pour la démocratie. Le remplacement du Cnesco, organisme indépendant dont la qualité des travaux est reconnue de tous, par un organe qui n'aurait plus pour mission d'évaluer les politiques éducatives et dont la majorité des membres seraient nommés par vous-même et par vos successeurs, monsieur le ministre, participe de la même logique. Un ministre qui voudrait regagner la confiance commencerait par entendre la contestation qui s'exprime depuis plusieurs semaines, il prendrait en compte les mobilisations, il écouterait les critiques, il traduirait les orientations données par le Président de la République à l'issue du grand débat- je pense par exemple à l'objectif de 24 élèves par classe, de la grande section

d'essence ultralibérale, qui sape les fondements de notre système scolaire. La confiance, c'est donner de la réalité à la promesse d'une école qui fait réussir le plus grand nombre et qui- enfin -réduit les inégalités. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors des assises de la maternelle, en mars 2018, le Président de la République affirmait : « Il y a toujours quelque chose d'éminemment politique au au sens le plus noble et le plus profond du terme, lorsqu'on parle [ ...] de l'éducation, parce que c'est là que l'on construit la société qu'on a à faire et qu'on veut voir ». Nous ne pouvons que souscrire à ce propos, tant l'école constitue le fondement même de notre société, le creuset de la République et de ses valeurs. Parce que l'éducation constitue justement un sujet politique, chacune des réformes entreprises en la matière provoque réactions et débats. Mais ce texte a suscité de réelles inquiétudes. Les polémiques actuelles s'inscrivent tout d'abord dans un contexte plus global : depuis le début du quinquennat, vous avez engagé de multiples réformes éducatives, détricotant les acquis de la loi de refondation de l'école de 2013, épuisant l'ensemble des acteurs concernés, las de devoir appliquer de nouvelles dispositions alors même que les effets des précédentes n'ont encore été ni mesurés ni évalués. Alors qu'enseigner et apprendre nécessite du temps, les enseignants et les élèves sont les premiers affectés par ces changements à marche forcée. Dans le contexte de crise sociale et politique actuel, les enseignants ont tenté de faire entendre leur voix par de nouveaux modes de contestation, attirant désespérément votre attention sur la dégradation de leurs conditions de travail et de leur pouvoir d'achat, sur le manque de reconnaissance, sur les violences quotidiennes, sur leur désarroi face à leur incapacité à répondre aux besoins de leurs élèves, faute de moyens, et sur les difficultés prégnantes qu'ils rencontrent trop souvent avec leur hiérarchie. Hélas ! le présent texte n'apporte pas de réponse à ces cris d'alarme, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources humaines et le bien-être des personnels : aucune mesure visant à assurer le suivi psychologique et médical, aujourd'hui inexistant, Pourtant, la confiance et la bienveillance passent aussi par la responsabilité de l'employeur vis-à-vis de ses personnels, qui, je le rappelle, Au-delà du contexte général, le projet de loi en lui-même inquiète l'ensemble des acteurs : la méthode, dénuée de toute concertation, n'a pas permis de les associer à la rédaction du texte. Le recours aux ordonnances témoigne aussi d'une volonté de limiter le débat parlementaire. Vous conviendrez, monsieur le ministre, que la confiance ne peut nullement se décréter dans un article de loi, quand ce dernier suscite la défiance des principaux intéressés. En dépit des stéréotypes parfois véhiculés moquant leur corporatisme et leur résistance au changement, les enseignants ont en réalité toujours su adapter leur pédagogie aux évolutions de la société. Faites-leur confiance ! Si ce projet de loi visait initialement à traduire dans le droit la volonté du Président de la République d'abaisser l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans, force est de constater qu'il engage, en réalité, de nombreux et profonds changements de notre système éducatif, tout en en taisant la plupart des aspects concrets et opérationnels, dont il eût pourtant été intéressant et nécessaire de débattre. Jugé trop disparate, décrit comme un « fourre-tout législatif », il interroge sur sa cohérence propre et son articulation avec l'ensemble de votre politique éducative. En réalité, il apparaît clairement que vous engagez, depuis deux ans, une vaste transformation du système éducatif : une éducation marquée par l'autonomie des établissements, par la concurrence, par l'évaluation, et d'une école à deux vitesses. Le projet de société que vous y dessinez, profondément ancré dans une conception libérale, ne répond ni aux enjeux du système éducatif ni aux difficultés auxquelles notre société est aujourd'hui exposée avec une acuité sans précédent. Une question demeure : quelle plus-value apporte ce projet de loi au système éducatif, à la réussite de nos élèves et à la lutte contre les inégalités ? Monsieur le ministre, la confiance, celle qui lie nos concitoyens et l'institution scolaire, ne pourra être restaurée que lorsque l'école de la République disposera des moyens nécessaires et suffisants pour remplir sa mission essentielle garantir à chacun, et en particulier aux plus vulnérables, la possibilité de se hisser au meilleur de ses capacités, en enrayant tous les déterminismes, pour qu'ils aient l'envie et le plaisir d'aller à l'école.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous commençons ce jour l'examen du projet de loi pour une école de la confiance. La multiplicité et la diversité des sollicitations dont nous avons pu faire l'objet témoignent des préoccupations profondes de la communauté éducative, des élus locaux et des parents d'élèves. Certaines objections ont pu être formulées à l'aune d'inquiétudes qui ne sont pas nécessairement fondées- nous le reconnaissons volontiers, monsieur le ministre. Toutefois, ce phénomène, particulièrement prégnant pour ce texte, n'est peut-être pas étranger à l'insuffisance du dialogue et de la concertation engagés en amont de son élaboration. Ce projet de réforme est venu se heurter aux attentes des Français, qui demeurent intactes, six années après la promulgation de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Les études PISA successives montrent, depuis près de deux décennies, une évolution assez alarmante du système éducatif français. Une des tendances les plus préoccupantes réside sans doute

Notre collègue Françoise Laborde et notre rapporteur, Max Brisson, ont commis, l'an passé, un rapport sur l'attractivité du métier d'enseignant que vous avez vous-même qualifié, monsieur le ministre, « d'inspirant La reprise, par notre commission, de plusieurs de leurs préconisations, comme l'inscription de l'obligation de formation continue de tous les professeurs, vient donc très opportunément enrichir ce texte. Notre groupe, au travers du dispositif de préprofessionnalisation ouvert aux assistants d'éducation, salue une disposition qui a vocation à familiariser les futurs enseignants avec le terrain scolaire. Toutefois, nous demeurons soucieux d'encadrer finement ce dispositif, afin que son objet ne soit pas détourné. Le RDSE se félicite également des nouvelles dispositions tendant à ce que l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire à 3 ans ne pèse pas, outre mesure, sur les budgets communaux. Notre groupe s'est particulièrement mobilisé sur ce point. Par deux fois, lors des questions au gouvernement, je vous ai interrogé, monsieur le ministre, sur l'accompagnement financier que le Gouvernement entendait mettre en oeuvre du fait de l'obligation nouvelle qui sera faite aux communes de participer au fonctionnement des écoles maternelles privées sous contrat. Le raisonnement de l'exécutif consistant à dire « qui faisait quoi avant ? » ou « qui engagera des dépenses nouvelles ? » ne pouvait nous satisfaire. La Haute Assemblée a donc voulu poser un principe équitable, les deux tiers des communes concernées accompagnant déjà, de manière facultative, l'enseignement maternel privé sous contrat. Nous nous sommes donc attachés à ce que toutes les communes soient soutenues financièrement et pas uniquement celles qui engagent une dépense nouvelle. Je profite de l'évocation de ce point pour attirer votre attention sur une autre réforme scolaire en vue qui ne sera, là encore, pas sans conséquence financière pour nos communes. Il s'agit de l'extension aux grandes sections de maternelle du dispositif de dédoublement des classes en réseau d'éducation prioritaire, ainsi que du plafonnement à 24 élèves, à l'horizon 2022, des effectifs, hors « REP », des classes de grande section de maternelle, de CP et de CE1. L'ouverture de 10 000 classes supplémentaires n'aura en effet rien d'anodin pour nos collectivités, qu'il s'agisse de locaux ou de personnels dédiés. Le 30 avril dernier, j'ai voulu vous interroger sur ce sujet.

Le renforcement de l'apprentissage des fondamentaux est primordial, et nous l'appelons, avec constance, de nos voeux. Mais nos élus locaux ne veulent plus d'un État dont les réformes qu'il lance engagent surtout les autres, et ce sans consultation préalable. En dépit d'une dynamique démographique tendant à réduire les effectifs du premier degré, personne ici ne se risquerait à dire que nos écoles publiques souffrent très majoritairement de surdimensionnement chronique. Là encore, le Sénat est dans son rôle lorsqu'il appelle le Gouvernement à la plus grande vigilance sur ce point. Monsieur le ministre, nous souscrivons pleinement à l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire, même si sa portée, en termes d'accueil, demeurera toute relative dans la grande majorité des territoires français. Les sénateurs du RDSE ont souhaité apporter des aménagements à cette mesure, afin de mieux prendre en compte le rythme biologique des élèves en petite section ou de pérenniser des structures existantes, comme les jardins d'enfants, qui ont toujours donné pleine satisfaction. Sur proposition de notre collègue Jean-Yves Roux, les membres de notre groupe ont, en outre, obtenu l'inscription du principe d'un accueil de l'enfant au plus près de son domicile. Le présent projet de loi introduit également une obligation de formation pour les jeunes de 16 ans à 18 ans. Nous comprenons la démarche qui tend à poser le principe d'une obligation d'éducation et de formation de 3 ans à 18 ans, mais les conditions dans lesquelles a été introduite cette disposition, par voie d'amendement et sans étude d'impact, révèlent une impréparation certaine et réduiront vraisemblablement cette mesure à l'état de symbole. Les conditions d'exercice et d'encadrement de l'instruction en famille ont aussi fait l'objet d'une attention particulière de notre commission. Notre groupe, notamment par le biais des propositions portées par notre collègue Nathalie Delattre, continuera de veiller à ce que ce recours, souvent précieux, ne soit pas dévoyé. Le RDSE partage aussi pleinement la position de la commission qui a conduit à la suppression de l'article portant création d'établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux. Sur la forme, le législateur ne saurait valider un dispositif aussi considérable sans étude ou évaluation préalables. Sur le fond, les craintes suscitées sont craintes suscitées sont nombreuses, notamment en termes de concentration scolaire « forcée » en zone rurale. Alors que la notion de proximité est revenue au coeur du débat public, cette disposition paraît bien inopportune. concerne la création du Conseil d'évaluation de l'école, le groupe du RDSE aurait plutôt souhaité voir évoluer les prérogatives du Cnesco. Nous adhérons toutefois aux aménagements apportés par notre rapporteur pour renforcer l'indépendance et la pluralité de la future structure. Le RDSE aurait également été partisan d'une poursuite de l'expérimentation du dispositif des PIAL, et de son évaluation, avant de procéder à un déploiement plus important. L'école inclusive représente un défi majeur.

Les sénateurs de notre groupe ont enfin porté et soutenu la suppression de la demande de réforme par ordonnances de la carte académique. En effet, au regard des annonces récentes du Gouvernement, une telle disposition ne paraît plus adaptée.

sans se soucier des incidences financières sur les collectivités locales et sur les maires ? Les lois se succèdent, et ne se ressemblent pas : Berthoin, Haby, Savary, Jospin, Fillon ... Parlerons-nous de la loi Blanquer dans quelques années ? L'histoire nous le dira.

alors même que 58 % de directeurs d'école déclaraient, en 2018, avoir subi des bousculades, des insultes, voire des agressions. L'article 3 crée une obligation de formation jusqu'à 18 ans. N'est-ce pas encore un engagement de communication du Président de la République, alors que le retour en formation ou à une formation professionnelle existait déjà ?

que mon groupe, de supprimer cet article et de le réécrire avec toute la sécurité demandée et souhaitée. Déjà, en 2019, à l'Assemblée nationale, un rapport montrait l'intérêt de cette école. Déjà, Frédéric Reiss parlait de regroupement. Déjà, Yves Durand parlait de la mise en amélioration

des collectivités territoriales et de la communauté éducative, d'un établissement correspondant à l'école du socle et nommé « établissement public local d'enseignement du socle commun

Il nous faut rappeler que le collège et les écoles qui composent cet établissement peuvent être implantés sur plusieurs sites, et non sur un site unique dans le collège, comme on a pu l'entendre.

Oscar Wilde disait que « le seul moyen de se débarrasser d'une tentation, c'est d'y céder ». Avec ce projet de loi, monsieur le ministre, vous venez conforter cette maxime. N'aviez-vous pas annoncé, en début de quinquennat, qu'il n'y aurait pas de loi Blanquer ? La vie politique est ainsi faite Quelle est, à l'origine, la motivation principale de ce texte ? Sans aucun doute, celle de concrétiser la promesse du candidat Macron de porter à 3 ans l'âge de l'instruction obligatoire. Au nom de quoi, de quel principe ? Permettez-moi de m'inscrire totalement en faux par rapport à l'argumentaire, souvent développé, selon lequel, avec cette mesure, notre pays disposera de la plus forte précocité en Europe en termes d'instruction. Je Je considère que l'on ne prend pas des mesures politiques pour battre des records, tout particulièrement dans le domaine si sensible de l'éducation nationale ... Tout acteur de la communauté éducative pourra convenir, avec un minimum d'objectivité, que le rythme d'un enfant de 3 ans n'est pas systématiquement adapté à une journée d'école qui démarre souvent dès sept heures trente, pour finir parfois après dix-huit heures. J'ai ainsi proposé un amendement, adopté en commission, qui vise à déroger à cette règle pour les plus jeunes, à l'issue d'une concertation entre parents, directeurs et équipes éducatives. Par ailleurs, il me semble important de redire que la cellule familiale doit rester le premier éducateur de l'enfant. J'ajoute que, au lieu de porter spécifiquement les efforts sur les départements qui se signalent par une singularité- ils ont été évoqués voilà quelques instants -, on généralise à l'ensemble du territoire national, sans anticiper sur les conséquences,

Bien sûr, comme tout texte touchant à l'école, celui-ci n'a pas manqué d'hystériser le débat public, à l'image de la mobilisation contre l'article 6 , qui créait les établissements publics locaux d'enseignement Parents d'élèves, personnels de l'éducation, enseignants et directeurs d'école ont beaucoup critiqué cette mesure avec, il faut bien le dire, des interprétations parfois malheureuses, et pas toujours objectives, tant s'en faut. Toutefois, comme trop souvent malheureusement, la méthode d'introduction de cette mesure n'était pas la bonne. Aussi, les membres de la commission de la culture et notre rapporteur Max Brisson, dont je salue le travail de grande qualité, ont-ils su entendre su entendre les craintes. Dans un souci d'apaisement, nous avons fait le choix de supprimer l'article 6 , au motif qu'il risquait, pour paraphraser mon collègue Jacques Grosperrin, de « constituer un cheval de Troie pour des regroupements non désirés Il faut néanmoins laisser une large place à l'expérimentation, car nous savons que ce dispositif correspond, localement, à des besoins réels. Poursuivant en quelque sorte la même logique que pour l'instruction obligatoire à 3 ans, le Gouvernement a introduit, à l'Assemblée nationale, l'obligation d'instruction jusqu'à 18 ans. Là encore, je m'interroge sur les effets visés. L'article 3 dispose que tout individu devra être inscrit dans un établissement scolaire, ou en formation, ou en emploi. Mais où serait-il donc si tel n'était pas le cas ? J'ai la nette impression que nous connaissons tous la réponse et que le mal profond auquel elle fait référence nécessite bien davantage qu'une mesure cosmétique de contrainte, qu'il sera bien difficile de faire respecter dans certains quartiers, surtout en confiant la mission de contrôle aux petits bras musclés de nos missions locales. Absolument ! Quitte à dépenser 100 millions d'euros en année pleine, j'aurais tellement aimé qu'on les destine à des dispositifs qui ont fait leurs preuves, comme les écoles de la deuxième chance. chance. Par ailleurs, le rôle des futurs assistants d'éducation doit absolument être précisé dans ce texte, pour éviter, là encore, des suspicions de mesures simplement budgétaires. La pratique, aux côtés d'un professionnel expérimenté, doit être encouragée, mais elle ne peut se transformer en système de remplacement. remplacement. L'article 1donne généralement le ton d'un texte. Comme vous le savez, monsieur le ministre, cet article est ici à l'origine de bien des manifestations hostiles de la part du corps enseignant. Il faut reconnaître que la notion d'exemplarité est tellement sujette à interprétation tellement imprécise, qu'elle ne peut que susciter la défiance, ce qui est l'exact contraire de l'objectif annoncé par le titre de ce projet de loi. Il me semble que le terme de « neutralité » serait plus adéquat. Je vous proposerai également, mes chers collègues,

Ce respect dû aux enseignants devrait aussi être un principe que les organisations syndicales s'appliquent à elles-mêmes, en commençant par respecter les directives de leur ministre de tutelle, qui a indiqué clairement que l'écriture inclusive, par exemple, n'était pas acceptable. Sur ce point, je suis en parfait accord avec vous, monsieur le ministre. L'essentiel est le retour aux fondamentaux sur le vocabulaire et la grammaire.

Pour nous en rendre compte, nous devons regarder l'ensemble des changements réalisés sous ce gouvernement. La réforme du lycée, dont l'application renforcera les inégalités territoriales, a succédé à la mise en place problématique de Parcoursup et à une nouvelle organisation des rythmes scolaires à la carte. À cela s'ajoutent les suppressions de postes, plus nombreuses chaque année, alors que les 60 000 postes créés lors du quinquennat précédent avaient tout juste permis de compenser les suppressions effectuées sous la présidence de

Vous mettez à mal l'école, notre École- avec un grand E -, sans concertation avec celles et ceux- élus, notamment ruraux, parents, communauté éducative -qui vivent l'école au quotidien. Et tout cela, sans aucune évaluation de ce qui a été fait précédemment. Vous empilez une nouvelle loi Blanquer, alors que ce dont notre école a besoin aujourd'hui, c'est d'un frein au train incessant des réformes, pour prendre enfin le temps de mettre en place ce qui existe. Ce projet de loi est un catalogue, un patchwork de mesures qui vont affecter structurellement notre système éducatif. Si son fonctionnement est encore à améliorer, vous proposez, avec ce texte, non pas une vision politique de l'éducation, mais une vision comptable qui consiste à trouver des professeurs qui coûteront le moins cher possible, au détriment de la qualité des conditions d'apprentissage des enfants, des enfants, ou à réduire le nombre de directeurs et de directrices d'école, alors qu'ils, et elles, sont le lien indispensable entre les différents membres de la communauté éducative. Quelques dispositions peuvent, certes, aller dans le bon sens. Je pense au meilleur contrôle de l'instruction en famille ou à l'instruction obligatoire dès 3 ans, une mesure que nous défendons depuis plusieurs années. Mais même sur ces points, nos craintes persistent, car ces réformes ne doivent pas être mises en oeuvre au détriment des communes. Nous nous inquiétons également de la suppression du Cnesco au profit d'un conseil constitué de membres désignés en grande partie par le ministère. L'indépendance des instances d'évaluation est cruciale, autant pour l'impartialité de ses évaluations que pour l'engagement pédagogique du corps enseignant. Ce texte met aussi en place une mise en concurrence des établissements. Ainsi, sous couvert d'expérimentation, la répartition des heures d'enseignement par matière pourra différer d'un établissement à l'autre. C'est aussi, comme je le soulignais, des choix purement comptables. Je pense, par exemple, au fait de confier des missions d'enseignement, de façon tout à fait prématurée, aux assistants d'éducation, dès la L2, lorsqu'ils, ou elles, se destinent à l'enseignement, afin de compenser les suppressions de postes et de réaliser des économies. Quant à l'article 6 , point dur du texte, dont nous saluons le retrait à l'unanimité par la commission, nous ne saurions accepter de le réintégrer sous une rédaction peut-être plus habile, mais aux conséquences tout aussi néfastes pour les territoires et le service public de l'éducation.

n'entraînera pas la fermeture de classes -mettront gravement à mal le lien social que l'école maintient dans les communes rurales. Ce n'est pas notre modèle d'une politique éducative de proximité.

À gauche, l'école de la République doit être un lieu d'émancipation individuelle et collective, un lieu d'acquisition des savoirs et des connaissances culturelles et, pour toutes et tous les élèves, un lieu de formation de citoyens éclairés, responsables, libres. Cela ne peut se faire sans le personnel enseignant ni la communauté éducative sur lesquels vous faites planer une suspicion injuste au travers de l'article 1. Ce sont eux qui font face, en première ligne, aux difficultés scolaires du quotidien. Ils ont besoin de reconnaissance, de respect, d'une revalorisation de leur métier, de moyens humains et financiers. tout simplement besoin de confiance. Monsieur le ministre, vos choix politiques sont cohérents et clairs. Ce texte n'est pas sans rappeler les attaques incessantes dont notre système scolaire a été victime entre 2007 et 2012- un affaiblissement grave auquel vous aviez d'ailleurs pris part. Vous faites l'éloge de l'employabilité comme objectif premier de l'école,

je crois aux forces de l'esprit. Là où il est, Jules Ferry ne peut qu'être interpellé par le nom de votre projet de loi, monsieur le ministre : « Pour une école de la confiance ». La plupart d'entre nous, ici, sont les filles et les fils de l'école de la République, cette République qui, dans les années 1880, a sonné le carillon de la plus heureuse et de la plus silencieuse des révolutions. En offrant à tous les enfants l'accès au savoir, qui était jusqu'alors avant tout réservé aux catégories les plus aisées, elle leur permettait aussi d'espérer une progression sociale par la réussite scolaire, les mérites de chacun Alors que le suffrage universel a établi l'égalité des droits, c'est l'instruction publique qui fut la servante consacrée de l'égalité des chances. École, méritocratie et République sont donc intimement liées dans notre histoire et notre mémoire collective. Or, depuis plusieurs décennies, la confiance entre les Français et leur école est fissurée. Preuve éclatante du malaise scolaire : l'exode massif d'élèves de l'école publique vers le privé. Personne ne peut croire que cette « fuite des cerveaux » soit due à une quelconque fièvre religieuse. Dans l'esprit de bien des parents, l'école privée d'aujourd'hui est tout simplement l'école publique d'hier, ... N'importe quoi ! ... celle où l'autorité du maître, le respect que les élèves lui témoignent et la valorisation des efforts étaient des fondements incontestables et incontestés. Bien des enseignants doutent, eux aussi. Mal payé, peu considéré, le professorat n'attire plus, tandis que des mouvements comme « les stylos rouges » ou « PasDeVague » illustrent cette grogne qui monte au sein de l'éducation nationale. Oui, monsieur le ministre, il faut rebâtir ce socle de confiance indispensable pour que notre école retrouve sérénité et efficacité. Malheureusement, à la lecture du projet de loi déposé à l'Assemblée nationale, quelle déception, tant, loin d'une grande loi sur l'école, révélait un bouquet fourre-tout, sans harmonie, sans ambition, sans vision. Quant à la mesure emblématique, l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans, déjà en vigueur quasiment partout dans l'Hexagone- je n'oublie pas, cela dit, nos amis de Mayotte et de la Guyane

qu'il s'agisse de la décapitation du « père » et de la « mère » dans les documents administratifs ou de la création des obscurs établissements publics des savoirs fondamentaux. Si certains se sont saisis du flou de cet article 6 pour agiter les peurs et cristalliser les ressentiments, force est de constater que l'on a rarement vu texte plus mal écrit. « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément »- ces vers de l'de Nicolas Boileau sont à méditer.

qui a permis d'améliorer le texte. Je pense notamment aux amendements relatifs à l'école inclusive, même s'il reste, en la matière, beaucoup à faire, au retour au bon sens et à la sagesse concernant les jardins d'enfants, à l'affirmation du rôle et de l'autorité des directeurs d'école. Espérons que l'examen qui s'ouvre sera fertile et que l'attitude positive et constructive de la Haute Assemblée, jamais démentie, recevra l'écoute souhaitée de la part du ministère. L'école de la République a besoin d'un nouveau souffle

soumettrai -que les intentions qui sont derrière ce projet de loi sont tout simplement les intentions affichées. Autrement dit, il n'y a aucune autre intention que celle qui est affichée. Vous avez le droit d'être contre ces intentions ; mais si vous ne voulez pas contribuer à alimenter cette société du soupçon

Puisqu'il a été fait référence à Jules Ferry, faisons un peu d'histoire. Si une grande loi se mesure au nombre

Je félicite mon collègue rapporteur Max Brisson de son travail de qualité ; il rappelle que le respect est d'abord dû par les élèves et leurs familles aux professeurs, à l'ensemble des personnels et à l'institution scolaire. Le second principe qui me paraît fondamental pour instaurer la confiance est la proximité. C'est pourquoi j'ai tenu, avec bon nombre de mes collègues, à ce que nous ne généralisions pas l'expérimentation relative aux établissements publics des savoirs fondamentaux, qui pourraient porter atteinte à ce principe.

serait menacée- ces écoles comptant peu de classes, un regroupement de classes peut signifier une fermeture d'école. J'ai eu la chance d'aller à l'école de mon village, qui était une école à classe unique.

Vous êtes venu dans le Puy-de-Dôme en 2018 ; vous avez pu y constater la réalité d'une école primaire riche de ses maîtres et la vitalité d'un collège rural.

Pourtant, il s'agit d'un texte dont l'adoption bouleverserait en profondeur le fonctionnement du système éducatif, mais sans aucune certitude de progrès. Compliqué, il l'est aussi dans son esprit. Ce texte, qui se veut ambitieux, doit être, selon vos propres mots, le socle d'une école qui inspire confiance et qui crée de la confiance en permettant la réussite et l'épanouissement de l'élève dès le début de sa vie ». Pourtant, monsieur le ministre, ce texte fait l'unanimité contre lui, chez les enseignants en particulier, au sein de la communauté éducative en général, et même chez un très grand nombre de parents d'élèves ! Si l'ambition du texte est de ramener de la confiance dans le monde enseignant, par ailleurs particulièrement en souffrance, la tâche est ardue,

J'ai bien conscience que cette question devrait être traitée dans le prochain projet de loi de réforme de la fonction publique. Mais j'insiste sur le fait

La méfiance à tous les échelons finit par affecter négativement notre modèle social et la perception que chacun peut avoir de l'État providence. En 2012, ces mêmes auteurs, ainsi que d'autres économistes, prolongent l'analyse et expliquent les causes de cette défiance, notamment l'obsession française pour les classements, l'inertie liée à son fonctionnement pyramidal et la fragmentation horizontale qui en résulte. L'école n'échappe pas à ce constat. sondage réalisé par l'IFOP, en 2018, 65 % des Français considèrent que le système scolaire ne garantit plus l'égalité des chances. Autrement dit, la promesse républicaine attachée à l'école apparaît comme une illusion.

en instillant implicitement une forme de défiance à l'encontre des personnels de l'éducation nationale, en particulier des professeurs, et ce dès l'article 1 du projet de loi Tel n'était peut-être pas votre objectif initial, mais tel a été le résultat, comme vous avez pu le constater. On pourrait d'ailleurs s'interroger sur la portée normative de ces dispositions, comme l'a fait le Conseil d'État dans son avis- cela a été dit. En d'autres termes, l'intention est louable, mais il n'est nul besoin de la loi pour répéter la loi le ministre, vous avez choisi de réaffirmer le devoir de réserve des personnels de la communauté éducative, et, au premier chef, celui des enseignants. Ce faisant, vous suscitez le doute, l'incompréhension

? Le lien de confiance qui unit les élèves et leurs familles au service public de l'éducation suppose de l'écoute et de l'apaisement. Pour cette raison, il nous semble plus que nécessaire de retirer cet article du projet de loi.

! Vous vous êtes approprié des concepts que vos prédécesseurs- je pense en particulier à Vincent Peillon

disposition qui n'a aucune valeur normative, qui existe déjà dans le code de l'éducation : bien entendu, les professeurs doivent être exemplaires,

toutes les études européennes montrent une corrélation entre le niveau de rémunération et le niveau de réussite scolaire.

d'une école tournée vers le monde, qui offre aux enfants la possibilité de s'épanouir et de prétendre à un avenir prometteur. Une école de la confiance ne doit pas inspirer de craintes, de doutes, de suspicions sur les intentions qu'elle affiche- je

Une école de la confiance implique aussi une reconnaissance de la spécificité et des besoins de chaque territoire. Il en est ainsi, notamment, de nos écoles rurales, qui pâtissent souvent de regroupements imposés. Il ne faut pas non plus oublier le travail accompli par les élus locaux de ces territoires, qui ne ménagent pas leurs efforts pour préserver leurs écoles, attirer des familles et faire vivre ainsi leurs villages. Notre ruralité souffre déjà trop de la disparition de multiples services publics. Il ne faut pas y ajouter la disparition de nos écoles, souvent liée aux fermetures de classes. La réduction du nombre de contrats aidés, dont ceux d'auxiliaires de vie scolaire, pourtant nécessaires, a été un coup dur porté aux services offerts aux enfants dans nos territoires ruraux. Cette mesure porte atteinte aux efforts de redynamisation de ces territoires oubliés de la République.

Il faut bien en parler : nous savons tous ici que les territoires ruraux, qui ne sont pas classés en REP, souffrent de la fermeture de classes et d'un taux d'encadrement dégradé, parce que l'on prend en compte des ratios peu adaptés aux écoles et établissements scolaires avec de faibles effectifs.

quelle politique vous comptez mener pour faciliter les relations, hors de tout conflit, entre familles et équipes enseignantes. Les parents font en effet partie de la communauté éducative. Il faut réfléchir aux moyens

Sur la forme, le Conseil d'État s'est interrogé sur la portée normative de cet article. Il considère que, si ces dispositions expriment certaines des valeurs incontestables autour desquelles l'école républicaine est fondée, elles ne produisent par elles-mêmes aucun effet en droit et réitèrent des obligations générales qui découlent du statut des fonctionnaires comme de lois particulières assorties, le cas échéant, de sanctions pénales. De son côté, le Conseil constitutionnel rappelle que la loi a vocation à énoncer des règles et censure les dispositions manifestement dépourvues de toute portée normative. Sur le fond, après la suppression de la notion de « respect mutuel » en commission, cet article stigmatise plus encore les parents en insinuant que, par principe, ils ne respecteraient pas l'école à laquelle ils contribuent par leur parole et leur engagement. Nous, maires et anciens maires, savons

que le premier article d'une loi s'intitulant « pour une école de la confiance » vise à encadrer- parce que c'est de cela qu'il s'agit ! -la liberté d'expression des personnels de l'éducation nationale.

J'avais été frappée par le fait que ces enseignants victimes de violences, qui sont peut-être les mieux à même de réfléchir sur ce qui nous rassemble aujourd'hui, faisaient preuve d'une hauteur de vue exceptionnelle et avaient une confiance absolue dans l'éducation pour faire face à ces phénomènes. Je crois

rien n'est prévu en cas de non-respect des principes énoncés dans l'article par l'une des parties de la communauté éducative. Le problème des incivilités au sein de la communauté éducative est pourtant réel et recrudescent. J'ai été moi aussi vraiment

que le législateur a déjà prévu des dispositions dans le code de l'éducation : il s'agit de l'article L. 111-4, qui traite des relations entre les parents, les professeurs et les autres personnels. Néanmoins, comme je viens de le dire, une simple déclaration de principe ne permettra malheureusement pas de résoudre les nombreuses situations conflictuelles. Les termes employés dans le dispositif de l'article, comme celui d'« exemplarité », risquent même d'envenimer les relations et de faire peser la suspicion sur le comportement de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, sans qu'aucun outil concret ne permette de remédier aux comportements inappropriés des personnels ou des élèves et de leurs familles. Ces considérations nous conduisent à demander la suppression de cet article.

l'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui unit les élèves et leur famille au service public de l'éducation. »

implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire. » Le fait

verbales et parfois physiques de la part d'élèves ou de parents d'élèves. Oui, cet article accentue la protection que nous devons aux professeurs. C'est le sens de ce que nous proposons et l'intention visée par cette loi. Je suis très heureux de pouvoir clarifier devant vous

L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui unit les élèves et leur famille au service public de l'éducation.

comme des hussards noirs. Sveltes ; sévères ; sanglés. Sérieux, et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. [ ...] Ces hussards noirs

Max Brisson de l'avoir réintroduit. En effet, l'autorité est indispensable pour qu'un professeur puisse transmettre le savoir. L'autorité implique aussi le respect. Quant à l'exemplarité, notre débat sur ce sujet est peut-être quelque peu byzantin.

Le scrutin est ouvert.

Le présent amendement vise donc à affirmer l'autorité des enseignants dans les établissements scolaires, condition nécessaire à l'exercice de la profession et à l'accomplissement de leurs missions au sein de l'école de la République. Je propose une rédaction différente de l'alinéa 2 de l'article 1, en

d'exemplarité et d'engagement, comme si ce n'était pas déjà le cas ! Par conséquent, nous préférons supprimer ces termes litigieux et prévoir que le seul lien de confiance entre les personnels de la communauté éducative, les élèves et leurs familles entraînera un respect mutuel et permettra la bonne marche du service public de l'éducation.

par la référence à la loi de 1983 sur la liberté d'expression des fonctionnaires, qu'aucun changement n'est prévu pour elle. Inutile d'alerter et de susciter la défiance de la communauté éducative alors que cette disposition « ne produit par elle-même aucun effet de droit et réitère des obligations générales », comme l'a relevé le Conseil d'État dans son avis sur le projet le projet de loi. Cet amendement ne tend pas à modifier la rédaction de la deuxième phrase, qui réaffirme que la relation entre l'élève et l'enseignant est une relation d'autorité, dans laquelle le respect est d'abord dû au personnel et à l'institution scolaire. Toutefois pour répondre complètement aux inquiétudes des enseignants, dans le cadre du mouvement « PasDeVague », une prise en charge plus large du phénomène est requise. Divers rapports ont préconisé l'installation d'un médiateur. Un véritable plan de lutte national contre les violences à l'école, annoncé par le Gouvernement, mais plusieurs fois ajourné, est nécessaire pour apporter des réponses concrètes et sortir des postures idéologiques. Nous restons vigilants quant au contenu et à la date de publication de ce plan, dont l'application est d'ores et déjà annoncée pour la rentrée prochaine. L'amendement n° 221 rectifié, présenté

abstraite et peut installer un climat de défiance vis-à-vis de cette dernière. Cet amendement vise à préciser que l'exemplarité attendue des enseignants s'entend plus précisément et plus particulièrement au regard

« doit unir » les élèves et leur famille au service public de l'éducation. Marc. Tout à l'heure, notre excellent collègue Philippe Dallier craignait que l'article 1 ne soit que déclamatoire. Je propose donc que le lien de confiance soit

De même que les partenaires des établissements d'enseignement et de l'éducation nationale participent de la communauté éducative, les personnels de l'éducation nationale participent utilement à la vie citoyenne grâce à leurs compétences propres. Plusieurs enseignants ont appelé l'attention des parlementaires sur des dispositions du présent projet de loi qu'ils estiment contestables. Le texte de ce projet de loi est public : lui appliquer une lecture critique participe des prérogatives des citoyens et ne contrevient pas en soi aux obligations des fonctionnaires. Pourtant, dans l'Hérault, un enseignant également adjoint au maire qui s'est exprimé publiquement pour appeler les sénateurs à exercer leur esprit critique sur le présent projet de loi a été convoqué par le directeur académique, qui l'aurait réprimandé. Il a reçu une lettre le rappelant à l'ordre. Si ce document n'est pas présenté par son auteur comme une sanction, son versement au dossier individuel de l'intéressé risque de nuire à ses évolutions de carrière et à ses demandes de mutation. Au-delà du grief, la démarche est de nature à intimider tous les membres de l'éducation nationale. Le présent amendement vise donc à préciser que l'engagement et l'exemplarité, que le présent article vise à inscrire dans le code de l'éducation, et qui font la richesse et la spécificité de l'apport des enseignants aux élèves, se mesurent aussi à l'aune de l'apport à la vie citoyenne

En outre, le respect dû par les élèves à leurs professeurs est remplacé par la mention d'un lien de respect entre les membres de la communauté éducative.

n° 221 rectifié, je partage pleinement l'intention de M. Piednoir : l'exigence d'exemplarité s'entend bien sûr au regard de l'obligation de neutralité des enseignants. Cette précision ne paraît toutefois pas utile : cette intention ressort clairement de nos travaux, sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire dans la loi. De surcroît, cette précision pourrait être réductrice l'exemplarité est plus large que l'obligation de neutralité. C'est d'ailleurs à l'occasion de violences sexuelles commises par un enseignement sur des mineurs en dehors du service que le Conseil d'État a affirmé

Comme tous les fonctionnaires, les enseignants sont soumis au devoir de réserve, dont les conditions sont définies par la jurisprudence administrative. Il s'agit d'un régime subtil et protecteur des agents, qui tient compte de leur rôle hiérarchique. C'est le corollaire de l'obligation de neutralité, qui ne se résume pas à la laïcité. Cet amendement tend à remettre en cause ce fragile équilibre.

malade. Les causes en sont multiples. Parmi ces facteurs, la perte de l'autorité du professeur en est probablement le symptôme le plus manifeste, suscitant une forte diminution de la reconnaissance sociale des professeurs. C'est ! La place privilégiée qu'ont occupée les enseignants dans la société reposait précisément sur la qualité de leurs connaissances et sur l'autorité qu'ils tiraient de leur mission de transmission. C'est certain ! Les multiples reformes engagée ces dernières années ont manifestement affaissé l'autorité des professeurs.

l'école ! La parole du professeur est de plus en plus « concurrencée » par l'envahissement du numérique. Or l'école devrait être préservée et être à l'abri de ce mouvement général de destitution du savoir et de déclassement du professeur.

mais il reprendra néanmoins le contenu des lois qui organisent le fonctionnement de notre école.

J'aimerais savoir si, comme cet enseignant de l'Hérault, il a été et réprimandé, et jusqu'où doit aller l'exemplarité d'un professeur de faculté ?

révérence. Nous sommes dans un état de droit, autrement dit, s'il y a le moindre problème dans la façon dont l'inspecteur d'académie a jugé le comportement de tel ou tel enseignant, la loi sera respectée. Il se

comme vous l'indiquez justement, du règlement intérieur des établissements. Pour ces raisons, je vous demande de retirer cet amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable. Quel est

L'objet de cet amendement est tout simplement d'en donner un commencement d'exécution. Les professeurs ne sont pas les égaux des élèves : ils incarnent l'autorité et l'ordre, tandis que les élèves sont dans une phase de formation et d'apprentissage- apprentissage des savoirs et du respect vis-à-vis des adultes. Se lever lorsqu'un professeur arrive, c'est un signe de courtoisie, de reconnaissance et de respect pour celui qui diffuse et transmet le savoir. Aujourd'hui, cette pratique est laissée à la discrétion des établissements et des professeurs elle doit être partout obligatoire, monsieur le ministre, et je ne puis croire que vous ne soyez pas d'accord avec ce principe de respect. Je vous demande de ne pas esquiver ce débat, car c'est une question importante. Monsieur le ministre, si vous considérez à juste titre que cette mesure réglementaire n'a pas sa place dans la loi, seriez-vous prêt à diffuser une circulaire- cela dépend de vous -pour inviter les établissements à inscrire cette disposition dans leur règlement intérieur ?

en prévoyant notamment la possibilité d'effectuer une retenue sur les allocations familiales versées aux parents d'élèves de moins de 16 ans. En effet, la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère a évalué, en mars 2018, le nombre d'élèves absentéistes à 250 000. Elle relève également que, de septembre 2017 à mai 2018, dans les établissements publics du second degré, quelque 5,6 % des élèves ont été absents, de façon non justifiée, demi-journées ou plus par mois, en moyenne. Ce taux d'absentéisme a crû en moyenne de 0,7 point pour l'ensemble des établissements par rapport à l'année 2016-2017, et le taux d'absentéisme moyen annuel est de 3,2 % dans les collèges, de 6,8 % dans les lycées d'enseignement général et technologique et de 18,3 % dans les lycées professionnels. En outre, l'absentéisme est plus élevé dans les établissements socialement défavorisés. Il s'agit donc d'une réalité tangible, qui impose aux pouvoirs publics de réagir. Le défaut d'assiduité des élèves influant nécessairement sur leurs résultats scolaires, il convient de ne pas laisser les jeunes obérer leurs chances d'avenir. L'amendement tend donc à faire de la responsabilisation des parents, éducateurs de leur enfant, un élément clé de la lutte contre l'absentéisme, au moyen d'un contrat de responsabilité parentale permettant de leur faire prendre conscience de la gravité de la situation. À cet égard, les parents bénéficient d'un accompagnement dans le cadre de ce contrat, et la complexité des situations individuelles est prise en compte. La sanction administrative se veut plus dissuasive que punitive. Elle est rendue nécessaire par l'insuffisance du dispositif mis en place au moment de la suppression de la loi dite Ciotti du 28 septembre 2010 par la loi du 31 janvier 2013, qui se limitait à renforcer le dialogue parents-établissements et à prévoir un personnel référent.

en 2013, visant à lutter contre l'absentéisme. Il a pour objet d'introduire un mécanisme de responsabilisation, fondé sur un contrat de responsabilité parentale, et de permettre, en dernier recours, une sanction par une retenue sur les allocations familiales.

dans le futur cette bonne relation entre les parents et l'école. Lorsque l'on parle d'école de la confiance, il est question de la confiance en eux des élèves, de la confiance qu'on leur donne dans le futur, mais aussi de la confiance entre tous les acteurs. On a beaucoup parlé de la confiance de l'institution envers ses professeurs et des professeurs envers l'institution, mais l'un des grands enjeux, c'est la confiance entre les parents et l'institution. À cet égard, la situation en France

la matière entre les parents et l'école. C'est pourquoi la coéducation est, à mes yeux, un bon concept : elle sous-tend qu'il existe une responsabilité partagée entre l'institution scolaire, entre l'école de la République et les parents,

l'article 371-1 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant », donc, notamment, l'éducation.

avoir. Certes, la coresponsabilisation des familles et des enseignants est une très bonne chose, mais cela ne suffit peut-être pas. Je suis totalement opposée à la suppression des allocations familiales,

seulement ont été rétablies, et dans 77 % des cas, l'enfant n'était pas retourné à l'école. Il est donc prouvé que cette mesure n'était pas efficace et dissuasive.

On risque à nouveau de diviser la famille, sans même d'ailleurs que la mesure ne produise une efficacité réelle ». Comme en 2014, chers collègues, je vous demande de nous retrouver sur des valeurs fondamentales, à savoir l'universalité des allocations familiales et la défense de la famille.

ils ne respectent pas une de leurs obligations prévues par le code civil au titre de l'autorité parentale. Des mesures d'assistance éducative sont possibles ; mais nous n'en avons pas les moyens.

Merci